La conférence des présidents a inscrit un débat sur le thème « Harcèlement scolaire : quel plan d'action pour des résultats concrets ?» à l'ordre du jour du mardi 11 avril 2023, à quatorze heures trente et le soir. À la demande du groupe Les Républicains, auteur de la demande d'inscription, ce débat aurait lieu sous forme d'une discussion générale. Il n'y a pas d'observation ? Il en est ainsi décidé. fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier est parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales. La parole est à Mme Françoise Gatel,

Ce vaste plan a déjà permis à la gendarmerie nationale non seulement de répondre présent lors de la crise sanitaire, mais également de modifier son paradigme opérationnel pour « aller vers » nos concitoyens. En matière d'effectifs, des efforts importants ont déjà été consentis lors du précédent quinquennat

Un tiers des 200 nouvelles brigades ainsi créées prendra la forme d'unités itinérantes, vouées à se déplacer dans les communes les plus éloignées des autres services publics de proximité. La création des brigades fixes permettra par ailleurs de réduire géographiquement la zone de compétence des brigades existantes, et donc d'alléger leur charge. Avec le déploiement de nouvelles capacités numériques, les gendarmes bénéficieront d'outils de travail qui permettront d'améliorer leur mobilité, de se rapprocher des usagers et d'optimiser le service. Les usagers pourront également contacter des gendarmes vingt-quatre sur vingt-quatre et sept jours sur sept grâce à différents portails numériques, parmi lesquels la brigade numérique, créée en 2018, qui rencontre un véritable succès auprès de nos concitoyens. L'optimisation du temps des gendarmes reste une préoccupation de la gendarmerie nationale. Elle expérimente dans plusieurs unités l'affectation de militaires du corps de soutien afin de décharger les gendarmes des tâches administratives. Cette démarche devrait monter en puissance. La parole

Elle est la seule BMR à compter deux spécialistes en réglementation transfrontalière- et pour cause ! -et deux analystes en fraude documentaire. Depuis sa création, cette unité a su développer une expertise certaine dans tout le Grand Ouest et des relations de confiance avec les élus et les habitants, tout en menant un travail partenarial avec de nombreux services, notamment sociaux.

s'ajouterait à d'autres restructurations préjudiciables au Calvados, comme celle du commissariat de la commune d'Hérouville-Saint-Clair à propos de laquelle j'ai déjà attiré l'attention du Gouvernement.

Parmi les mesures prises, je veux citer la création, le 1 janvier dernier, d'un nouvel office central spécialisé, l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim), rattaché à la police aux frontières (PAF). Par sa forte dimension interministérielle et ses capacités de pilotage opérationnel et stratégique, ce nouvel office va permettre de lutter plus efficacement contre les réseaux criminels de passeurs. Pour ce faire, il s'appuiera sur un réseau territorial- antennes et détachements -constitué à partir des actuelles BMR et de la PAF. Le réseau des BMR est donc amené à évoluer : une grande majorité des brigades deviendront des antennes ou des détachements de l'Oltim. La cartographie définitive de ce nouveau réseau territorial n'est pas encore arrêtée : nous y travaillons encore, avec nos services, pour trouver l'organisation territoriale la plus efficace et adaptée possible. Vous serez informée personnellement de la place qu'occupera dans ce dispositif l'actuelle BMR du Calvados. Sur le second point de votre question, la circonscription de sécurité publique de Caen, dont dépend Hérouville-Saint-Clair, compte en effet à ce jour un effectif opérationnel de 310 gradés et gardiens de la paix, alors qu'ils étaient 272 à la fin de de 2016. J'ajoute que 28 policiers adjoints sont affectés à cette circonscription de police. Quant au commissariat de secteur d'Hérouville-Saint-Clair, qui fait partie de cette dernière et qui bénéficie donc de ses moyens, il dispose en propre d'un effectif opérationnel de 17 gradés et gardiens de la paix ; il peut également s'appuyer sur 4 policiers adjoints.

sur l'existence de la décharge sauvage envahissant le fort militaire de la Redoute, propriété du ministère de l'intérieur. Cette décharge à ciel ouvert est située à proximité immédiate de l'Institut Gustave-Roussy, ainsi que du parc départemental des Hautes-Bruyères. Le contraste entre ces trois lieux est saisissant. Le premier est le théâtre d'un scandale sanitaire majeur, résultat d'une criminalité environnementale sur laquelle la justice s'est déjà prononcée. Depuis la période du confinement, ce sont près de 40 000 mètres cubes de déchets toxiques, soit environ 20 800 tonnes de gravats, en vrac ou ensachés, de plaques de fibrociment brisées, de carcasses d'électroménager, d'amiante, de plomb, de cyanure et de mercure qui jonchent le site, qui pénètrent les sols avec les eaux qui en découlent et qui aggravent dangereusement la qualité de l'air. Les amoncellements de matériaux culminent jusqu'à douze de mètres de hauteur et envahissent les espaces voisins. Le second site, l'Institut Gustave-Roussy, a vocation à devenir l'un des premiers pôles mondiaux de recherche et de traitement du cancer. En investissant 100 millions d'euros dans le Campus

est un espace de curiosité, de détente et de loisirs qui accueille 85 parcelles de jardins familiaux et de nombreux promeneurs. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous préciser le calendrier et les mesures prises par l'État pour procéder, dans les plus

? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Lafon, vous m'interrogez sur le cas d'un dépôt de déchets qui se trouve sur le territoire de la commune de Villejuif dans le Val-de-Marne. Tout d'abord, je souhaite être claire : il est inadmissible que nos paysages et nos espaces naturels ou urbanisés soient pollués par des déchets abandonnés ou stockés en toute illégalité. Qu'il s'agisse de dépôts illégaux ou de véritables décharges exploitées illégalement, ces amas de déchets non seulement sont de vrais dangers environnementaux et sanitaires, mais peuvent aussi, dans certains cas, mettre en danger nos concitoyens en cas d'incendie. Pour le cas particulier du site de la Redoute de Villejuif, le terrain a été occupé par la préfecture de police pour des activités de formation depuis la fin des années 1960. L'activité a cessé progressivement à partir des années 2000 et la préfecture de police a quitté le site en 2016. Entre 2020 et 2021, les bâtiments du fort de la Redoute ont été illégalement occupés et dégradés et des déchets se sont accumulés lors de cette occupation. Le Gouvernement est conscient de la situation et confirme que des études sont en cours pour la mise en oeuvre de mesures visant à l'évacuation des déchets présents. De manière générale, la résorption des dépôts sauvages de déchets ou de décharges illégales est un sujet sur lequel il faut passer à la à l'économie circulaire du 10 février 2020 a ainsi introduit des mesures pour agir à la racine sur les causes de la gestion illégale des déchets, financer certaines opérations de nettoyage, renforcer l'efficacité de la police des déchets, informer et former sur cette question. Le Gouvernement souhaite aller plus loin et donner à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable davantage d'outils pour combattre les activités illégales en matière de déchets. C'est bien le sens des orientations prioritaires données pour 2023 à l'inspection des installations classées sur ce sujet. La parole

Ce site accueillait il y a une dizaine d'années la Société industrielle de munitions et travaux, qui avait pour but de retraiter les explosifs, obus, torpilles et autres munitions de l'armée française. À la suite de la cessation d'activité de la société, le site est resté en l'état et regorge encore aujourd'hui d'armes instables, enterrées ou pas, en très grande quantité. Le pire est à craindre dans un lieu qui n'est même pas gardienné ! En 2015, le préfet prévoyait le placement de panneaux rappelant l'interdiction de pénétrer et informant du danger de mort autant dire une véritable publicité pour des personnes mal intentionnées ! Il faut savoir qu'à quelques mètres de ce terrain se trouvent un pipeline de pétrole brut et une usine de stockage de gaz. À ce stade, la menace d'une explosion en chaîne n'est donc pas à exclure. La nappe phréatique qui circule sous le site alimente tout le bassin de vie. Une opération de déminage a été menée du 19 au 23 avril 2021 au cours de laquelle 1 421 obus au phosphore ont été découverts. Depuis, plus rien ! Les déminages programmés n'ont pas été effectués. Le ministre de l'intérieur en faisait état dans une lettre qu'il a adressée à Mme la maire de Saint-Martin-de-Crau le 28 mars 2022 et dans laquelle il s'engageait « à étudier les solutions existantes pour assurer le traitement et la destruction de ces engins Un an après, votre étude devrait être enfin terminée- je l'espère, en tout cas ! -et vous devriez avoir la capacité d'agir pour dépolluer le site. Mais les élus locaux n'ont plus aucune réponse de la part

en 2016 pour l'enlèvement de la pollution restante. Ces opérations de dépollution, liées à la prise en compte et à la destruction de déchets pyrotechniques, dont les armées conservaient la responsabilité à la suite de la défaillance d'un opérateur privé, ont entraîné l'élimination de 120 tonnes d'engins de guerre. Aujourd'hui, la remise en état du terrain nécessite encore le traitement de plusieurs centaines de tonnes de munitions enterrées, dont environ 25 000 obus au phosphore. En surface, une caractérisation de danger doit encore être réalisée sur un amas de 350 tonnes de munitions diverses.

Aujourd'hui, de nombreux élus estiment que ces dispositions sont inadaptées et qu'elles posent de graves difficultés, notamment au moment où les marges de manoeuvre financières de nos collectivités locales se réduisent. Historiquement, le modèle d'investissement des collectivités dans la construction d'une gendarmerie permettait de ne pas faire peser l'accueil d'un casernement sur leurs charges de fonctionnement. Les nouveaux référentiels de sécurité établis par la gendarmerie nationale, la réglementation relative à l'isolation thermique et l'inflation engendrent une augmentation substantielle des dépenses que les communes doivent supporter. En Mayenne, la commune d'Évron s'est engagée aux côtés de l'État dans la construction d'une nouvelle caserne et de seize logements répondant aux normes environnementales et de qualité de vie au travail- un engagement local fort et légitime et légitime pour nos gendarmes. Mais le bilan prévisionnel de ce projet fait apparaître une perte importante pour la commune, de l'ordre de 100 000 euros par an. En effet, le budget est estimé à plus de 5 millions d'euros et il manque 1 million d'euros de financement, hors frais d'entretien, pour que l'équilibre financier soit respecté.

ruraux. La parole est à Mme la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Chevrollier, l'immobilier constitue le coeur du système d'arme de la gendarmerie nationale et occupe une part importante des projets à venir dans le cadre de la Lopmi. Au vu des difficultés financières rencontrées par la commune d'Évron, un ajustement des prescriptions attendues en termes de sécurisation de l'emprise et de l'ouvrage est en cours d'étude. ailleurs, des précisions seront apportées à la collectivité afin qu'elle puisse actualiser son plan de financement sur la base du programme fonctionnel désormais stabilisé, en intégrant le montant de la subvention d'État qui pourra être sollicitée en cours de chantier ainsi que le montant prévisible du loyer qui sera arrêté à la livraison. En outre, des financements complémentaires pourront utilement être recherchés, tant auprès de la préfecture que d'autres collectivités. Enfin, en application de la nouvelle réglementation sur les baux, le loyer- après une période invariable de neuf ans -sera révisé triennalement, selon la variation des indices de l'Insee qui prennent notamment en compte l'inflation, et cela jusqu'au terme de la vingt-septième année de location. Au regard de ces éléments, et si l'on prend en considération les garanties octroyées au maître d'ouvrage pendant les trois premiers baux de neuf ans, la chronique des différents flux financiers permettra de couvrir

La réforme de l'assurance récolte a pris effet au 1 janvier de cette année. Du fait de la répétition des événements calamiteux en raison du changement climatique, certains agriculteurs ont été sinistrés à plusieurs reprises au cours des dernières années. Tel est le cas des producteurs d'abricots des Baronnies qui, de 2017 à 2022, ont été chaque année victimes de gels ayant engendré des pertes importantes sur les récoltes, alors même qu'ils n'avaient connu aucun épisode similaire au cours des dix années précédentes. Pour ces agriculteurs pluri-sinistrés, la conséquence directe est que la référence historique de production, qui sert de base à tout calcul d'indemnisation, est très faible sur les cinq dernières moyenne triennale ou moyenne olympique. Ils se retrouvent donc sans protection possible pour 2023, puisqu'ils ne seraient que très faiblement couverts, que ce soit par un contrat d'assurance récolte ou par le fonds de solidarité nationale prévu pour les agriculteurs non assurés. En outre, il ne leur est plus possible d'augmenter leur capital garanti en évaluant leur production à un niveau de prix supérieur de plus de 20 % au prix de référence du barème national, car cela les priverait du bénéfice de la subvention politique agricole Cette situation inquiète non seulement les producteurs, mais aussi les organisations professionnelles et les services administratifs départementaux qui craignent, en cas de nouveaux aléas climatiques importants, de ne pouvoir déterminer les taux de perte de récolte demandés pour que les non-assurés puissent être indemnisés. Madame la ministre, ma question est simple : est-il possible de faire évoluer la réglementation en matière d'assurance récolte afin de prendre en compte les nombreux cas d'agriculteurs pluri-sinistrés au cours des dernières années ?

À long terme, le Gouvernement se fait le porte-voix de ces préoccupations relatives à la référence historique auprès des instances européennes. Dans certaines situations, l'augmentation de la fréquence des aléas climatiques peut conduire à ce que la référence à un potentiel de rendement historique entraîne une dégradation de la référence de production historique, quelle qu'en soit sa définition.

Pour autant, et pour tenir compte de l'évolution des coûts de production, les exploitants ont la possibilité de s'assurer à un prix allant jusqu'à 120 % de la valeur de ce barème tout en bénéficiant de garanties subventionnables. Enfin, les exploitants qui désireraient s'assurer à une valeur de prix plus élevée peuvent le faire sans perdre le bénéfice des aides à l'assurance en souscrivant à des garanties non subventionnables complémentaires proposées par les assureurs. La parole

Cette méthode intègre l'ensemble des surfaces en prairie, alors les éleveurs n'en gèrent qu'une partie. Le calcul du besoin de fourrage est ainsi fondé sur un indice mis en place il y a une vingtaine d'années, déconnecté des besoins actuels.

Madame la ministre, entendez-vous modifier les indices de calcul du déficit fourrager, afin que les éleveurs touchés par la sécheresse puissent à l'avenir bénéficier de l'indemnisation ? La

Ces dernières proviennent essentiellement du système indiciel utilisé dans le cadre du dispositif de l'assurance subventionnée des prairies. À l'occasion de la réforme de l'assurance récolte, Marc Fesneau a confirmé l'ambition de remettre en place un réseau de fermes de référence pour renforcer dans la durée la confiance de tous en assurant le suivi

toujours plus intenses et fréquents. L'investissement dans la formation à la prévention et à la gestion des risques climatiques, crucial pour faire face aux conséquences du changement climatique, sera traité au sein du pacte et de la loi d'orientation et d'avenir agricoles. La parole

nationale et de la jeunesse. Ma question porte sur la possible disparité du niveau de difficulté des épreuves du baccalauréat dans une même spécialité et sur la manière dont l'équité peut être assurée une fois l'inégalité constatée.

Pour cette raison au moins, il semblerait équitable que les élèves passent tous l'épreuve d'une même spécialité le même jour, sur un ou plusieurs sujets identiques.

niveau de difficulté. Madame la ministre, pour quelles raisons n'est-il pas possible d'imposer qu'une même épreuve, surtout s'agissant d'une spécialité à fort coefficient, soit organisée le même jour pour tous les élèves l'ayant choisie Je souhaite également savoir quels moyens de compensation sont disponibles et susceptibles d'être utilisés pour lisser les inégalités entre les candidats, en particulier alors qu'en mathématiques spécialisées, par exemple, une disparité de niveau, mais aussi de longueur de sujet, semble objectivement constatée entre l'épreuve de la veille et celle du lendemain ? La parole

possibles. Depuis la session 2022, première session pour laquelle les épreuves de terminale dans leur nouveau format ont pu être mises en oeuvre, l'organisation de l'examen

permet aux centres d'accueil collectif de mineurs de déroger à certains aspects du droit du travail, notamment sur le volet de la durée journalière de travail et sur la rémunération. Ce dispositif souple répond aux besoins quotidiens induits par les larges amplitudes horaires de ces centres, notamment

plan que vous présentiez l'an dernier aux assises de l'animation, vous annonciez, dans la mesure 24, que ces contrats d'engagement éducatifs seraient réservés à l'avenir « aux seuls accueils collectifs de mineurs avec hébergement Comme bien d'autres, le centre de loisirs Saint-Ferréol, situé à Bon-Encontre, près d'Agen, dans mon département du Lot-et-Garonne, est inquiet depuis cette annonce.

part, la suppression des CEE pour des structures telles que le centre de loisirs de Bon-Encontre réduirait des deux tiers les capacités d'accueil, dégradant ainsi considérablement la qualité du service sur le territoire. Madame la ministre, face à tant d'inquiétudes, quelles réponses êtes-vous en mesure d'apporter à tous ces centres d'accueil collectif qui font la richesse de nos territoires et qui, désormais, redoutent une fermeture inéluctable ?

le Gouvernement est attaché au maintien et au développement dans nos territoires d'une offre de loisirs de qualité au bénéfice du plus grand nombre de jeunes. Cet objectif ne peut se concrétiser sans une action forte en faveur de l'attractivité des métiers de l'animation. des engagements pris durant les assises de l'animation, qui ont été lancées en octobre dernier par Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel,

adaptées. La réflexion engagée autour du contrat d'engagement éducatif s'inscrit bien dans cet objectif. En effet, la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Les métiers de l'animation connaissent un déficit d'attractivité, qui donne lieu à des pénuries de personnel. Personne ne peut donc se satisfaire du. Comme vous le savez, le contrat d'engagement éducatif est un contrat dérogatoire au droit commun, notamment en matière de durée de travail, de repos et de rémunération. Il semble adapté aux conditions d'organisation des accueils collectifs de mineurs avec hébergement. question de l'utilisation de ce contrat dans les accueils sans hébergement doit être posée. Le comité de filière Animation, installé durant les assises, a notamment pour mission de formuler des propositions de « définir une trajectoire pour revaloriser significativement le minimum légal de la rémunération et réserver ce contrat aux seuls accueils collectifs de mineurs avec hébergement ». Dans ce cadre, les différents acteurs du secteur, en particulier les organisations représentatives des employeurs et des salariés, devront se prononcer sur le sujet. L'objectif est donc double : assurer la viabilité économique du secteur et offrir de réelles perspectives professionnelles aux animateurs. Un bilan intermédiaire est prévu le 14 juillet prochain.

les fermetures de classes et de postes sont toujours plus nombreuses, s'accentuant d'année en année : déjà 1 493 écoles ont été supprimées en cinq ans. Après ces baisses successives, vous avez également annoncé la suppression de 1 500 postes dans les écoles pour la rentrée de 2023. Paris est particulièrement touché : le rectorat a décidé la suppression, dès la prochaine rentrée scolaire, de 182 postes d'enseignants dans les collèges et lycées et la fermeture de 178 classes dans les écoles primaires. Cette baisse continuera pendant les trois prochaines années, avec une diminution de 600 classes au total. Nous avons bien conscience de la baisse démographique dans la capitale.

Une étude de l'OCDE publiée en 2022 montre que la France est l'un des pays comptant un nombre d'élèves par classe parmi les plus élevés. Inversons cette tendance ! Le nombre d'enfants par enseignant joue un rôle sur la qualité des apprentissages et constitue l'une des explications de notre mauvaise position dans les évaluations internationales du niveau scolaire. En parallèle, les écoles privées de Paris se voient doter de moyens importants, alors qu'elles ne jouent pas le jeu de la mixité.

après une baisse démographique de 300 000 élèves ces cinq dernières années, 500 000 élèves de moins sont attendus d'ici à 2027 à l'échelle nationale.

public, soit une baisse de 20 % des effectifs. Cette tendance s'est accélérée ces dernières années. Une baisse de 3 178 élèves dans les établissements du premier degré est prévue pour la rentrée scolaire prochaine. L'académie de Paris détient le meilleur taux d'encadrement de France métropolitaine, après la Corse,

élèves à Paris pour une moyenne nationale de 17,8. Toutes les classes qui ont été dédoublées en grande section, en CP et en CE1 dans les écoles relevant de l'éducation prioritaire le resteront ; celles qui doivent l'être le seront. Aucune de ces classes ne verra ses effectifs dépasser Je crois que nombre d'académies envient la situation de Paris. Les conditions d'enseignement y sont excellentes, les faits parlent d'eux-mêmes. Dans le second degré, une baisse démographique de près de 2 % est attendue entre les rentrées scolaires 2022 et 2023. Là encore, les taux d'encadrement y sont bien plus favorables que dans le reste de la France. Par ailleurs, s'il y avait besoin de le rappeler, le maillage en établissements scolaires de la capitale est tel que chacun des élèves peut y accéder sans difficulté. Vous le voyez, monsieur le sénateur, l'académie de Paris est pleinement mobilisée afin que tous les élèves, tant dans le premier degré que dans le second, et tous les

la saison estivale se profile, mais les piscines des collectivités, des hôtels et des campings, particulièrement fréquentées dans mon département de l'Ardèche, vont-elles pouvoir ouvrir ? En effet, la pénurie de maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) demeure. La Fédération française de natation estime ainsi à 5 000 le nombre de postes vacants, autant de professionnels qui manqueront pour la sécurité des baigneurs et pour l'enseignement de la natation.

sont recrutés, reste le problème de la fidélisation des maîtres-nageurs sauveteurs. Au-delà de 2023, l'été 2024 fait craindre aux collectivités des difficultés encore plus grandes pour la surveillance de la baignade du fait de la mobilisation des CRS-MNS pour les jeux Olympiques. Les états généraux de l'encadrement et de la surveillance dans la filière aquatique, organisés le 10 février dernier, ont permis d'échanger et d'avancer, notamment sur les évolutions réglementaires, sur l'accès aux formations ou encore sur l'augmentation du nombre de certifications permettant d'obtenir le titre de MNS. la ministre, vous aviez annoncé le lancement d'une grande campagne de communication et de promotion pour encourager les vocations en amont de la saison estivale. Nous sommes déjà début avril : qu'en est-il ?

fermées ? La parole est à Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Ventalon, la pénurie de maîtres-nageurs et ses conséquences en matière de difficultés de recrutement pour les collectivités, l'hôtellerie et les centres aquatiques sont des situations bien identifiées par la ministre des sports. Celle-ci a réuni, le 10 février dernier, les états généraux de l'encadrement et de la surveillance dans la filière aquatique, afin de poser les bases d'un plan d'action. Ce dernier s'articule autour de la réglementation, de la formation, des conditions de travail et de la valorisation du métier. Il a aussi permis de préciser les échéances pour répondre à la situation d'urgence de la prochaine saison estivale. Ce plan prévoit une évolution réglementaire avant les prochaines vacances scolaires pour pour permettre aux collectivités et aux entreprises de recourir plus facilement aux titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), qui pourraient dorénavant exercer leur mission de surveillant sauveteur en autonomie dans tous les contextes de baignade, qu'elle soit gratuite ou payante. Ce plan fixe aussi des objectifs ambitieux en matière de formation, comme le déploiement de l'apprentissage dans le secteur privé ou dans la fonction publique territoriale et le développement d'une offre de formation continue

autour de l'attractivité des métiers de la fonction publique, dans le cadre du plan Accès, carrières et rémunérations, auront des effets sur l'attractivité de la profession de maître-nageur sauveteur, exercée à 80 % dans la fonction publique territoriale. En outre, je tiens à évoquer le lancement d'une campagne de communication nationale afin de promouvoir ce métier essentiel pour l'apprentissage

font trop peu souvent l'objet de poursuites, encore moins de condamnations. Les décisions de classement sans suite sont trop souvent la règle sans que la raison en soit communiquée et encore moins expliquée aux élus. Pourtant, la loi prévoit depuis 2021, sur l'initiative du Sénat, l'obligation non seulement d'informer, mais aussi de motiver le classement. Les maires vivent cette situation comme un manque de considération et une défiance à leur égard, d'autant que la voie judiciaire est bien souvent la seule qui permette de sanctionner les infractions dans des domaines relevant de leurs compétences, notamment en matière d'urbanisme. En novembre dernier, le garde des sceaux indiquait que « le dialogue avec les élus est désormais une priorité des procureurs ». Il est bien difficile de mesurer sur le terrain les résultats de cette annonce, car il n'existe aucun suivi de ces plaintes et signalements. Je demande Je demande depuis plusieurs années la mise en place d'outils permettant une transparence vis-à-vis des maires et une vision globale de la réalité des suites données à leurs plaintes et signalements. À une réponse à ma question écrite sur le sujet, il m'a été indiqué que « le ministère de la justice travaille à la mise en place d'applicatifs visant à faciliter, d'une part, le recueil de signalements et, d'autre part, le suivi de ces procédures ». J'aimerais donc savoir, madame la secrétaire d'État, où en est la mise en oeuvre de ces applicatifs de suivi et, au-delà, ce que le Gouvernement compte faire pour améliorer la prise en compte, le suivi et l'information des élus en ce domaine.

le ministère de la justice est pleinement engagé dans la lutte contre la délinquance du quotidien. Les maires, en tant que premiers relais de la République dans les territoires, sont des interlocuteurs privilégiés des parquets, le ministre de la justice l'a rappelé à plusieurs reprises. Au-delà des instructions fermes délivrées, le ministère de la justice a souhaité mettre à disposition des juridictions, à brève échéance, des outils permettant de renforcer concrètement leur action. C'est pourquoi, depuis le mois de février 2022, les services du ministère travaillent au développement d'un applicatif visant à assurer le suivi des politiques pénales prioritaires visées par les instructions que le garde des sceaux délivre régulièrement. Cet outil de suivi des politiques pénales prioritaires a justement vocation à permettre aux parquets d'assurer un suivi précis des situations référencées à ce titre. C'est évidemment le cas des infractions commises au préjudice des élus, tout comme des infractions signalées par ces derniers dans le cadre de la justice de proximité. Cet outil permettra, par le biais d'alertes automatiques, d'améliorer significativement le partage de l'information. Son déploiement à l'automne est d'abord, évidemment, centré sur le suivi des violences intrafamiliales. Il est ensuite axé prioritairement sur le suivi des atteintes aux forces de sécurité intérieure et aux élus. Ces fonctionnalités devraient être ouvertes d'ici à la fin de l'année 2023. Enfin, les services du ministère ont également développé la plateforme InfoParquet qui permet non seulement d'assurer un retour automatique sur les suites données à leurs signalements, mais également de doter les parquets d'un outil permettant de mesurer l'évolution du nombre de signalements dans un domaine particulier.

fin des recettes publicitaires, restrictions budgétaires, suppression de la redevance, restructuration administrative, plan de départs ... Voilà quelques semaines, un projet de fusion de France 3 et France Bleu a fuité. La note des directions de France Télévisions et de Radio France est très claire : « création d'une marque unique, mise en oeuvre d'un projet éditorial commun, rationalisation des implantations, création de directions uniques et développement de la polyvalence au sein des équipes ». Cette annonce a eu l'effet d'une bombe. Elle est ressentie par les personnels comme du mépris à l'égard du nécessaire dialogue social et comme une nouvelle attaque contre leurs missions et leurs compétences. Ils craignent, à juste titre, un plan social à peine dissimulé et une perte de qualité des émissions proposées au public. L'inquiétude est d'autant plus grande que les rapprochements intervenus ces derniers temps n'ont pas suscité l'adhésion, loin de là.

Quelle est la vision du Gouvernement concernant l'audiovisuel public et, plus précisément, le devenir de France Bleu et France 3 ? Où est passé l'engagement pris par la ministre de la culture au moment de la suppression de la redevance d'associer « le Parlement et les entreprises de l'audiovisuel public » à la définition des nouveaux contrats d'objectifs et de moyens (COM) adossés à une trajectoire de dotation pluriannuelle avec

En se transformant ces dernières années et en multipliant les coopérations, il s'est renforcé et imposé comme le premier média des Français en radio comme en télévision. Son développement numérique s'est accéléré. Le média global Franceinfo est devenu le premier site d'information en ligne de notre pays et sa couverture quotidienne a doublé en cinq ans ! Il s'agit bien d'un projet de coopération, le plus abouti de l'audiovisuel public. France 3 et France Bleu ont également commencé à unir leurs forces avec le déploiement des matinales filmées et le lancement d'une offre numérique commune, « ici », par France 3 et France Bleu. La ministre de la culture travaille avec les entreprises pour consolider et renforcer cette dynamique, qui portera ses fruits dans les prochains contrats d'objectifs et de moyens. Des pistes sont en cours d'expertise. La proximité constituera à n'en pas douter l'une des priorités priorités de ces COM. Toutes les enquêtes le montrent : les Français attendent davantage de proximité dans l'information, les programmes et les sujets traités. Leur défiance croissante à l'égard des médias traduit aussi un sentiment d'éloignement et le besoin que les médias soient plus proches de leur vie locale. Les coopérations entre France 3 et France Bleu ont vocation à être poursuivies et amplifiées. Il ne s'agit évidemment pas d'amoindrir une offre plus indispensable que jamais, mais bien de la renforcer. Elle doit gagner en puissance et en visibilité, notamment en ligne, et offrir une couverture toujours plus riche de la vie locale. Il est important que ces projets, s'ils devaient prospérer, se fassent dans le respect du dialogue social, en concertation avec les salariés et les organisations syndicales.

porte sur la réforme en cours de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Le champ des garanties prévoyance et les moyens que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre pour soutenir ces garanties protectrices pour tous - titulaires, contractuels, actifs et retraités - sont en train d'être arbitrés.

La réflexion sur le volet prévoyance peine pourtant à aboutir, notamment pour les personnels de l'État, où aucune construction de couverture cofinancée par l'employeur n'est aujourd'hui imposée par le cadre légal. La prévoyance risque donc fortement de devenir secondaire dans la réforme en cours, ce qui laisserait les agents dépourvus de garanties, alors qu'ils ont cotisé pendant de nombreuses années. De plus, pour les personnels territoriaux, les niveaux de couverture, corrélés aux aides financières des collectivités, risquent d'être inaccessibles pour les personnels aux plus bas revenus. Pour les hospitaliers, durement touchés, la prévoyance n'est toujours pas abordée. Qu'en est-il des discussions et réflexions au sein du ministère de la fonction publique ? Surtout, quelles garanties pouvez-vous donner aujourd'hui ? Il paraît urgent

afin de favoriser et d'améliorer la couverture sociale complémentaire des agents de la fonction publique. Avec cette ordonnance, l'employeur public a pris ses responsabilités- il est important de le souligner. Les employeurs publics sont en effet désormais tenus de financer au moins 50 % de leur complémentaire santé. Cette ordonnance permet également une participation de l'employeur à des contrats de prévoyance couvrant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès. Cette obligation s'applique bien aux trois versants de la fonction publique, tout en tenant compte des points de départ différents et des spécificités. La question de la protection sociale pose également celle de la prévoyance, qui est au coeur des négociations que mène actuellement le ministère de la transformation et de la fonction publiques avec les organisations syndicales. Celles-ci

améliorer les revenus de remplacement qu'ils servent - c'est ce qu'on appelle les garanties statutaires ou l'auto-assurance - ou recourir à des contrats de protection sociale complémentaire. De la même façon, des négociations se poursuivent dans la fonction publique territoriale et s'engageront dans la fonction publique hospitalière. D'ici à l'été, le ministère de la transformation et de la fonction publiques réunira les employeurs publics et les organisations syndicales des trois versants, afin de faire un premier bilan de la mise en oeuvre, par les employeurs, de l'ordonnance « protection sociale complémentaire ». La parole est

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, ma question porte sur l'application du dispositif d'emploi-retraite pour les élus locaux cessant leur activité professionnelle principale. Pour bénéficier du cumul emploi-retraite, ces élus sont dans l'obligation de liquider l'ensemble des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires auprès desquels ils cotisent. Cette situation place de fait l'exercice du mandat d'élu comme une activité donnant lieu à l'application du dispositif encadrant le cumul emploi-retraite, lorsque la personne concernée cesse son activité professionnelle principale, comme l'impose l'application des dispositifs prévus par le code de la sécurité sociale, dans la rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014. Une telle situation ne permet pas à l'élu de poursuivre une activité professionnelle principale au titre de l'emploi-retraite, sauf à engager les mesures susceptibles d'entraîner la liquidation de son régime de retraite auprès de l'Ircantec,

est dans l'obligation soit de démissionner de son mandat soit de renoncer à ses indemnités, pour répondre à l'obligation de liquidation de l'ensemble des régimes de retraite obligatoires obligatoires auprès desquels il cotise. Madame la secrétaire d'État, je souhaite savoir si le Gouvernement envisage de prendre les mesures réglementaires nécessaires pour que la cotisation auprès de l'Ircantec, en raison de l'exercice d'un mandat, ne fasse pas obstacle à la possibilité d'exercer une activité dans le cadre du dispositif d'emploi-retraite.

et la justice du système de retraites a harmonisé les règles de cumul d'emploi-retraite applicables au sein des différents régimes de retraite. Plus précisément, la loi a introduit le principe de cessation d'activité pour pouvoir liquider sa retraite et de non-constitution de droits nouveaux en cas de reprise d'activité. Le législateur a également clarifié le statut des mandats électifs au regard de ces nouvelles règles. Afin de ne pas décourager l'exercice d'un mandat local à la retraite, les règles du cumul ne font pas obstacle à la perception d'indemnités de fonction. Les élus ne sont donc pas obligés d'interrompre leur activité au moment où ils liquident leur retraite et peuvent continuer à percevoir leurs indemnités de fonction, ainsi qu'une pension. Ils bénéficient par ailleurs d'une mesure dérogatoire concernant le cumul emploi-retraite au titre de leur régime complémentaire obligatoire. Celle-ci leur permet de se constituer de nouveaux droits à retraite Ircantec. Ces droits ouverts les empêchent néanmoins d'accéder aux dispositifs de cumul d'emploi-retraite dit intégral. S'agissant des avocats, ils relèvent d'un régime de retraite de base distinct du régime général, lequel ne prévoit pas la possibilité de reprendre ou poursuivre une activité dans le cadre d'un cumul emploi-retraite plafonné. Seul le cumul emploi-retraite intégral leur est ouvert. Néanmoins, les modalités d'application de la création de droits nouveaux pour tous les assurés en cumul emploi-retraite prévues dans le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 devraient résoudre cette difficulté.

permettent de déterminer les concours financiers de l'État, au premier rang desquels la dotation globale de fonctionnement. En outre, 350 textes réglementaires font référence aux chiffres de population légale, dans de nombreux domaines : nombre d'élus au conseil municipal, détermination du mode de scrutin, ouverture de pharmacies ou réglementation sur l'hébergement d'urgence. Or il s'avère, de l'avis des maires comme des associations d'élus, que la méthode actuelle est particulièrement défavorable aux communes qui connaissent un accroissement de population, comme c'est le cas de plusieurs d'entre elles dans mon département de Seine-et-Marne. En effet, les effets de l'augmentation de la population ne sont pris en compte que plusieurs années après l'arrivée des nouveaux habitants sur la commune. Sont en cause le décalage entre la date de recensement et son entrée en vigueur, mais également un effet de lissage sur cinq ans, qui retarde la prise en compte de l'augmentation de la population. Les communes, de leur côté, doivent, dès l'arrivée des nouveaux habitants, engager des travaux pour agrandir l'école, créer de nouvelles routes, construire un gymnase et réaliser tous les autres investissements nécessaires pour garantir une bonne proportion de services publics. Elles doivent faire face aux nouvelles dépenses tout de suite, sans bénéficier des recettes qui leur reviennent. Autre sujet connexe, de nombreux territoires font état de défaillances notables dans les modalités de recensement, avec la non-prise en compte des portes closes, le phénomène de multi-location ou la suroccupation de logements, ce qui aboutit au même problème de différentiel entre les statistiques, qui déterminent les dotations, et la réalité du terrain. Madame la ministre, il paraît indispensable d'améliorer le dispositif actuel, pour mieux appuyer l'effort des communes qui accueillent de nouveaux habitants. Je souhaite savoir si vous envisagez une évolution de la méthode de calcul des populations légales pour mettre fin à ce décalage ou,, un mécanisme permettant de le compenser. je vous remercie le recensement de la population a été réformé en 2002 par la loi du 27 février relative à la démocratie de proximité. Depuis cette date, les chiffres de population d'une commune sont actualisés chaque année. Il n'est plus nécessaire d'attendre les résultats d'un recensement général. Les informations collectées sont ramenées à une même date pour toutes les communes, afin d'assurer l'égalité de traitement et de permettre une bonne fiabilité des données. Cette nouvelle procédure traite à égalité l'ensemble des communes, puisque c'est l'année médiane du cycle des recensements qui est retenue. Il n'est pas concevable qu'une commune reçoive une dotation calculée sur des chiffres plus anciens ou plus récents, du simple fait de sa taille ou en vertu du hasard ayant fixé la date du recensement. Les événements qui affectent positivement ou négativement la démographie d'une commune sont effectivement pris en compte avec un décalage de trois ans dans toutes les communes. Vous avez raison, cette méthode peut être défavorable aux communes qui connaissent une forte croissance de leur population. Mais elle est favorable à celles qui connaissent une dynamique inverse : en 2022, 43 % des communes ont vu leur dotation forfaitaire diminuer du fait d'une baisse de leur population. Or les deux types de communes doivent être traités de la même façon. Le recensement de la population fait l'objet d'une évaluation permanente, lors de laquelle il peut être proposé des modifications. C'est sans doute dans ce cadre que le débat pourrait être porté, si vous le souhaitez.

des nappes phréatiques sont à un niveau jugé inquiétant, la bataille de l'eau est à nos portes. Nous devons nous y préparer sans attendre. Pour cela, il est indispensable d'accompagner les communes et les intercommunalités dans la gestion de cette ressource autrefois abondante et bon marché qu'est l'eau. Trois axes m'apparaissent essentiels. Le premier est naturellement d'ordre financier, puisque 40 % du réseau a plus de 50 ans et que 20 % de l'eau se perd avant d'arriver au robinet. Les annonces présidentielles sont-elles à la hauteur des énormes besoins ? Avons-nous la garantie que

Nous sommes d'ailleurs revenus, voilà quelques jours, dans cet hémicycle, sur le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement, afin de donner davantage de souplesse aux municipalités. nous avons agi, au-delà de nos appels répétés sur ce retour nécessaire, dans la continuité du rapport du Sénat de novembre dernier intitulé, qui préconise notamment de décentraliser davantage la décision publique sur l'eau et de faire confiance aux échelons locaux. le troisième axe est de refuser et de combattre tout dogmatisme dans la gestion de l'eau et de sa rareté, loin d'une vision écologique rétrograde, incarnée par un extrémisme dangereux, comme nous avons pu le voir à Sainte-Soline ou ailleurs. Madame la secrétaire d'État, cette bataille se fera avec les élus locaux ou ne se gagnera pas.

le changement climatique a des impacts d'ores et déjà visibles sur le cycle de l'eau. La résilience de nos territoires est une priorité du Gouvernement. Ce sujet est au coeur des travaux de planification écologique portés par la Première ministre. Le plan Eau, en particulier, a été annoncé par le Président de la République le 30 mars En 2022, en anticipation de la sécheresse, 100 millions d'euros des agences de l'eau ont été dégagés en urgence, notamment pour engager des travaux de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable. à la sécheresse hivernale que nous rencontrons actuellement, cet effort a été renouvelé en 2023. La gouvernance de l'eau repose sur l'implication des collectivités et de leurs groupements pour porter la maîtrise d'ouvrage des opérations. L'échelon intercommunal a été choisi par le législateur pour remédier aux difficultés sanitaires, économiques et écologiques engendrées par l'émiettement des services d'eau et d'assainissement sur l'ensemble du territoire.

Les élus locaux sont encouragés à définir dans ces Sage les priorités d'usage de la ressource en eau et la répartition, sur leur territoire, Par ailleurs, des moyens supplémentaires sont apportés pour soutenir les collectivités les plus en difficulté. Face aux investissements importants pour réduire les fuites et sécuriser l'alimentation en eau potable, 180 millions d'euros par an, seront dédiées au petit cycle de l'eau et conditionnées à une amélioration durable de la gestion de l'eau de leur patrimoine. Le plan Eau renforce de manière inédite les capacités d'intervention des agences de l'eau, qui sont les principaux financeurs de la politique de l'eau aux côtés des collectivités.

par exemple le bornage, tandis que les seconds peuvent exécuter tous les travaux topographiques n'ayant pas d'incidence foncière. Pourtant, cette distinction est manifestement d'un autre temps, la technique topographique n'étant plus celle de 1946, de sorte que les opérations de bornage- monopole des géomètres-experts -sont bien moins complexes que les opérations topographiques. Ce monopole passéiste entraîne des conséquences

5 000 logements en copropriété. Outre son anachronisme, une telle décision serait totalement inopportune en termes d'efficience économique ». Madame la secrétaire d'État, avez-vous l'intention de mettre un terme à ce monopole ?

la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts reconnaît à cette profession un monopole sur la délimitation des biens fonciers. En France, la propriété est un droit constitutionnel. En réservant aux géomètres-experts la réalisation des études et des travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers, le législateur a entendu garantir la protection de la propriété foncière, en confiant sa délimitation à des professionnels spécialement qualifiés et présentant toutes les garanties que la loi impose. Si le progrès technique a facilité la réalisation des opérations de délimitation foncière, le professionnel engage cependant sa responsabilité sur ces prestations. Dans son avis de 2018, l'Autorité de la concurrence n'a pas remis en cause le bien-fondé du monopole. Toutefois, elle a recommandé de préciser la définition légale de ce monopole en matière de délimitation de la propriété foncière, en établissant notamment une liste qui définirait précisément les prestations qui relèvent du monopole et celles qui sont dans le champ concurrentiel. À cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 2022 conclut en particulier que la réalisation des plans annexés aux actes de division foncière relèverait du monopole des géomètres-experts. Un tel plan, dès lors qu'il est visé et annexé aux actes de copropriété, peut en effet contribuer à la délimitation foncière. L'Autorité de la concurrence a été de nouveau saisie par la Chambre syndicale nationale des géomètres-topographes. Le Gouvernement attend ses conclusions avant de statuer. La profession compte 1 878 professionnels. Les conditions d'accès à la profession ont été profondément assouplies par le biais du diplôme délivré par le Gouvernement. Pour faciliter encore l'accès à la profession pour les géomètres-topographes,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis 2012, l'usine de fabrication d'engrais Yara, située à Montoir-de-Bretagne, en Loire-Atlantique, ne cesse d'inquiéter.

Son bilan en matière de pollution atmosphérique est tout aussi sinistre. En 2020, Yara a rejeté plus de 200 tonnes de poussières, principalement constituées de particules fines. Dans l'agglomération nazairienne, le nombre d'hospitalisations pour affections respiratoires est plus élevé de 39 % à la moyenne nationale chez les moins de 18 ans. Un tel constat est insupportable Alertées, les autorités ont réagi. Cependant, malgré les nombreux arrêtés préfectoraux de liquidation d'astreintes ainsi que son intégration dans le plan national de vigilance renforcée du ministère de la transition écologique, l'entreprise refuse toujours de se mettre aux normes. Pire encore, interrogé lors du salon de l'agriculture cette année, le PDG de Yara France estimait être en mesure de demander à l'État une dérogation concernant les rejets atmosphériques Face à cette attitude inacceptable et qui n'a que trop duré, quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement ? Il y a urgence : ce comportement arrogant doit enfin cesser ! La parole

l'usine Yara située à Montoir-de-Bretagne fait l'objet de constats persistants de non-conformité depuis plusieurs années de la part de l'inspection des installations classées, notamment en matière de rejets atmosphériques et aqueux. La pression mise par les services de l'État a permis d'aboutir à des avancées majeures sur ce site, en particulier pour la prévention des risques accidentels. Cependant, l'exploitant doit encore mettre en conformité ses installations pour le traitement des rejets atmosphériques et celui des eaux industrielles et pluviales. Compte tenu de ces constats, ce site a été placé en vigilance renforcée dès juillet 2021. La société Yara a élaboré un plan de mise en conformité comportant des mesures concrètes, quantifiables et vérifiables, qui doivent être mises en oeuvre selon un échéancier déterminé. L'avancement de la mise en oeuvre de ce plan fait l'objet d'un suivi très attentif de l'inspection des installations classées et peut être consulté sur le site internet du ministère. Une réunion avec l'exploitant a été organisée le 10 novembre 2022,

La société Yara fait également l'objet de sanctions administratives, avec des astreintes financières d'un montant total de plus de 200 000 euros pour les années 2020 et 2021.

Actuellement, 4,5 % seulement des emballages de boissons consommées et moins de 10 % des emballages en verre mis en marché sont réemployés. Pourtant, pour parvenir à nos objectifs, le réemploi est incontournable. Il s'agit d'un processus vertueux pour le climat

d'économies pour le consommateur. Les sondages montrent que 88 % des Français attendent la consigne ! Madame la secrétaire d'État, y a-t-il une volonté politique de faire avancer le réemploi des contenants et des emballages ? Quelles sont les mesures envisagées à cette

les objectifs sont d'atteindre 10 % d'emballages réemployés en 2027 et de réduire de moitié le nombre de bouteilles en plastique à usage unique d'ici à 2030. Pour accompagner le développement des solutions de réemploi des emballages, un nouveau fonds de financement de 50 millions d'euros par an sera mis en place dès cette année avec les éco-organismes de la filière des emballages ménagers. La loi anti-gaspillage permet également de mettre en place un dispositif de consigne des bouteilles pour le recyclage et le réemploi. C'est dans ce cadre fixé par la loi que s'inscrit la concertation que j'ai engagée et dont vous êtes partie prenante. Il s'agit d'approfondir les leviers qui permettront d'améliorer la collecte des emballages et de développer le réemploi. Les travaux portent, notamment, sur les synergies qui pourraient exister entre la consigne pour réemploi et la consigne pour recyclage. Le réemploi fait partie des travaux de concertation engagés,

sur la nécessité d'investir dans des infrastructures de transports. En Moselle, cette nécessité nous est particulièrement connue. En effet, tous les jours, ce sont près de 120 000 salariés qui traversent la frontière vers le Luxembourg le matin et le soir. Sur l'autoroute A31, reconnue comme l'une des plus chargées de France, voire d'Europe, transitent de 10 000 à 15 000 poids lourds et plus de 100 000 voitures chaque jour. Dans ce pays des frontières, il y a encore la possibilité de relancer des voies et des gares- à Hayange, à Nilvange, à Fontoy

la Moselle reste à quai alors qu'elle est la porte d'entrée du Benelux et des pays du nord de l'Europe dans l'Hexagone l'A31. Je pourrais aussi évoquer l'absolue nécessité d'entamer au plus vite les études et plus encore les travaux pour mettre en place un réseau express métropolitain, sorte de RER régional entre Nancy-Metz et Luxembourg, alors que le Grand-Duché annonce près de 300 000 travailleurs pendulaires français à l'horizon de 2050 et que l'actuel TER, malgré toute la bonne volonté de la région, de la SNCF et de ses agents, ne suffit déjà plus à assurer un service de qualité. Aujourd'hui, madame la secrétaire d'État, les habitants du nord de la Moselle, mais je sais que mon ami Olivier Jacquin partage les mêmes préoccupations que moi pour le nord de la Meurthe-et-Moselle, souffrent des bouchons permanents, de la pollution, des maladies que cela entraîne, de l'usure accélérée des routes, des dangers d'une circulation embolisée par des infrastructures inadaptées. Allez-vous entamer sans délai des études sur un réseau express métropolitain et sur la relance de voies ferrées et du fret ferroviaire dans le nord mosellan ? Allez-vous mettre ces questions en tête du sommaire de la prochaine conférence intergouvernementale avec le Luxembourg ? Allez-vous inscrire prioritairement des investissements en faveur des infrastructures ferrées en Lorraine

fait l'objet d'investissements importants pour répondre aux enjeux de mobilité transfrontalière en forte croissance. Comme vous le savez, il s'agit effectivement de créer un véritable service express métropolitain dans le cadre d'un protocole d'accord entre la France et le Luxembourg signé en 2018 et modifié en 2021, consacrant près de 440 millions à cette ligne à l'horizon de 2030, à parité entre les deux pays.

de répondre à la saturation de l'axe dès 2024. Je pense à l'allongement des quais de gare, au renforcement électrique, aux parkings-relais à Thionville et à Longwy ou au pôle d'échanges multimodal de Une seconde phase d'amélioration capacitaire a également été identifiée à l'horizon de 2030 grâce à l'augmentation de la puissance électrique disponible, à la reprise du plan de voies à Thionville, à des aménagements sur le noeud de Metz ou encore à la création de deux sas fret. Concernant les prochaines étapes, commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise pour le renforcement de la coopération transfrontalière, qui se tiendra le 17 avril prochain à Thionville, sera l'occasion d'un point d'avancement sur l'amélioration des conditions de mobilité des frontaliers. L'élaboration du volet mobilités 2023-2027 du CPER Grand Est sera également importante pour la poursuite des investissements sur le réseau ferré lorrain, au-delà du seul sillon mosellan. La parole

aéroport est disposé à relever les défis de la souveraineté économique, de la transition écologique et de la qualité de vie des habitants. Ses points forts sont nombreux : une des plus longues pistes d'atterrissage d'Europe, une capacité de 200 000 tonnes de fret par an, un accueil de tous types d'avions, sept jours sur sept, vingt-quatre Les atouts et les potentiels de développement économique sont prêts à être déployés, mais l'aide de l'État et des responsables économiques est indispensable ! Je sais que la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et votre collègue des transports sont mobilisés autour de Vatry et attentifs à ses possibilités de développement. Il s'agit déjà de diriger les flux de fret de notre pays vers Vatry plutôt que vers d'autres plateformes étrangères concurrentes. En plus d'un meilleur bilan carbone, cette relocalisation d'activités en France aura des bénéfices financiers et fiscaux. Si l'on cherche un troisième aéroport francilien, chacun fera des économies, car il est déjà construit : il existe et il est en Champagne ! Vatry constitue une véritable opportunité pour l'Île-de-France de désengorger ses trafics aéroportuaires et d'offrir à ses habitants une réduction des nuisances sonores. Vatry offre un panel de solutions et un équipement opérationnel, normé et certifié. Il fait déjà ses preuves ! Madame la secrétaire d'État, je vous demande une mobilisation forte et imminente

jugez utile. La parole est à Mme la secrétaire d'État. Madame la sénatrice Férat, depuis l'ouverture de l'aéroport de Châlons-Vatry au trafic commercial en 2000, celui-ci fait l'objet d'un soutien important des collectivités territoriales propriétaires du foncier et actionnaires de la société d'exploitation. L'État accompagne leurs efforts depuis l'origine et encourage, dès que cela est possible, le développement des vols de fret vers les aéroports régionaux, notamment Vatry. Le fret aérien international étant transporté en majorité dans la soute des avions de passagers, il se concentre naturellement dans les grands aéroports de correspondance. Durant la crise sanitaire, l'aéroport de Vatry a joué un rôle essentiel dans l'acheminement du matériel médical sur le territoire national. La direction générale de l'aviation civile a en effet autorisé, à titre dérogatoire et de façon innovante, le transport du fret en soute, mais sans passagers, notamment vers Vatry. L'aéroport est devenu le septième aéroport de fret en France en 2021. Toutefois, en 2022, la demande mondiale de fret aérien s'est affaiblie et les vols de passagers ont repris. Par ailleurs, le revenu moyen du fret a chuté brusquement. Dès lors, et malgré les efforts déployés, l'aéroport de Vatry s'est trouvé confronté à d'importantes incertitudes économiques. Des projets privés qui s'étaient manifestés ne se sont pas concrétisés, faute de financement. L'État accompagne activement et au mieux le développement de cette infrastructure régionale. En particulier, un « groupe contact » associant la direction générale de l'aviation civile, la préfecture, le conseil départemental et l'aéroport a été mis en place à la demande du ministre délégué chargé des transports, Clément Beaune,

2022, l'État lançait une enquête publique dans le cadre d'un projet d'implantation, actuellement soumis à autorisation environnementale, d'un centre de fabrication de matériaux alternatifs à base de mâchefers, sur le territoire de la commune du Bar-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes.

ainsi que les administrés. En effet, s'ils reconnaissent l'intérêt public d'une telle installation, laquelle contribuerait au retraitement des déchets, tous dénoncent, à juste titre, son impact environnemental. Ce projet pose deux difficultés majeures.

déficitaire. Seconde difficulté, ce projet engendrerait une pollution atmosphérique importante, avec une explosion du trafic, et le passage régulier et exponentiel de poids lourds de déchets. Madame la secrétaire d'État, alors que l'enquête publique a pris fin, qu'entend faire l'État pour ajourner ce projet face à autant de griefs mobilisés sur ce territoire ?

vous attirez mon attention sur l'implantation d'un centre de production de matériaux à base de mâchefers dans les Alpes-Maritimes, qui suscite l'inquiétude des riverains. Les mâchefers sont issus de la combustion de déchets ménagers. Ils sont généralement utilisés dans le secteur des travaux publics ou enfouis. L'entreprise MAT'ILD propose une nouvelle solution de valorisation de ces mâchefers en les incorporant à la fabrication de béton de granulats. Cette activité industrielle est soumise à une procédure d'autorisation préfectorale stricte. Un dossier de demande d'autorisation a été déposé en mars 2022 par le porteur de projet. Il a fait l'objet d'une enquête publique en décembre 2022. Les services du préfet m'ont fait savoir que les avis recueillis dans le cadre de cette enquête publique sont mitigés. Le commissaire enquêteur a, de son côté, émis un avis favorable sur ce projet. Ce dernier doit encore être présenté pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst). Ces consultations permettront également de formuler des recommandations pour mieux adapter et renforcer les mesures de prévention des pollutions. Le préfet prendra ensuite une décision sur ce projet en tenant compte de l'ensemble de ces avis et de ces recommandations. Si ce projet venait à être autorisé, je tiens à vous assurer que les services de l'État seront particulièrement vigilants à ce que les mesures de prévention des pollutions soient pleinement respectées. La parole

mise en place début janvier 2022 devait faciliter la mobilisation des crédits issus du Dife. Or de très nombreux dysfonctionnements et blocages ont été constatés : droits pour un élu que la plateforme ne retrouve pas, nom de jeune fille ou marital déclaré introuvable, différents problèmes de validation des données saisies, soucis de règlement des formations

Faute de réussir à finaliser leur démarche, ils ont été privés de leur possibilité de formation en 2022. Il serait donc juste qu'ils puissent conserver leurs droits en 2023.

Monsieur le sénateur Reichardt, depuis janvier 2022, les élus peuvent directement mobiliser leur droit individuel à la formation Mon compte élu, une plateforme numérique adossée à Mon compte formation dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations Cette plateforme permet de fluidifier le parcours des élus et de réduire les délais de traitement. Les élus peuvent désormais consulter le montant de leurs droits, comparer les offres de formation sur l'ensemble du territoire, s'inscrire à des formations et y participer quelques jours plus tard. Le Gouvernement est conscient que ces nouvelles modalités ont pu temporairement complexifier les démarches des élus, d'autant que face aux nombreuses fraudes et tentatives de fraudes sur la plateforme il a mis en place des mesures de sécurité renforcée afin de préserver les droits des utilisateurs. Un niveau supérieur de sécurité de France Connect a été déployé depuis le 25 octobre 2022. Pour tenir compte des difficultés engendrées par ces évolutions et du temps nécessaire à l'appropriation de la procédure par les élus, un projet d'arrêté en cours d'adoption prévoit de relever de 700 euros à 800 euros le plafond des droits pouvant être détenus afin de ne pas pénaliser les élus qui n'ont pas utilisé leurs droits en 2022. Cela permettra donc le report intégral des droits de 2022 sur 2023.

les zones de revitalisation rurale (ZRR), créées en 1995, concernent 17 662 communes et 15 % de la population française. Les ZRR sont une forme de reconnaissance de la différenciation territoriale, en faveur de la particularité des territoires ruraux. En Aveyron, 100 % des communes sont concernées par ce dispositif, qui permet de favoriser le développement local par des aides fiscales et sociales soutenant la création ou la reprise d'entreprise, les salariés et les professions libérales. Les aides et exonérations temporaires accordées aux entreprises des communes qui en bénéficient servent à l'attractivité des zones rurales, ce qui est essentiel. En effet, l'économie dans les espaces ruraux, en particulier dans les espaces peu denses et très peu denses, repose largement sur leur attractivité professionnelle et sur l'offre de services qui y est dispensée, adaptée à une population souvent vieillissante ou à destination des familles. Vous comprendrez donc, madame la secrétaire d'État, que la fin du dispositif au 31 décembre 2023 suscite de fortes craintes. J'insiste pour vous faire part de ma grande inquiétude concernant la situation en Aveyron si le dispositif venait à disparaître. Cette inquiétude provient d'abord d'une incompréhension tout à fait légitime des élus locaux : pourquoi ne pas maintenir ce dispositif qui fonctionne ? Cette inquiétude provient, ensuite, du flou qui entoure la trop longue période transitoire à propos de laquelle nous savons trop peu de choses.

le Gouvernement partage avec vous le constat que vous faites sur l'importance des zones de revitalisation rurale et la nécessité de les pérenniser. Il est particulièrement mobilisé pour garantir l'accès aux services publics à l'ensemble de la population. Ainsi, tous les Français se situent désormais à moins de trente minutes d'un espace France services pour bénéficier d'un accompagnement dans leurs démarches administratives. Ce dispositif marque le retour des services publics dans les territoires ; le Gouvernement vous affirme son intention de le pérenniser. Le dispositif ZRR prévoit notamment des aides à l'installation en ruralité pour les entreprises. Ces aides contribuent grandement à lutter contre le manque d'attractivité dont souffrent parfois nos territoires ruraux pour accueillir, mais aussi maintenir de nouvelles populations. Les ZRR sont au centre des politiques que nous menons à destination des ruralités. Depuis l'été 2022, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Dominique Faure,

Les mesures qui seront retenues feront l'objet d'une large concertation et d'un travail rigoureux avec les sénateurs. Elles seront intégrées à un plan plus large en faveur des ruralités afin d'apporter des solutions concrètes et adaptées à chaque territoire. La parole

Cette situation est en effet source d'instabilité pour les collectivités territoriales dont les dépenses d'investissement deviennent moins prévisibles. Pour les communes de taille modeste et porteuses d'importants projets d'aménagement,

le flash FCTVA du 30 janvier 2023 en provenance de la préfecture, j'ai appris que les comptes 2128 et 2312 ont été retirés de la liste sans aucun motif apparent. Je tiens à préciser que, si des subventions départementales ou régionales sont sollicitées, le plan de financement prend en compte l'apport budgétaire représenté par le futur FCTVA. Pour une collectivité modeste qui verrait certaines dépenses inéligibles, c'est donc la double peine : pas de FCTVA et pas de subvention majorée. ailleurs, la nature de certains comptes non admis dans le périmètre FCTVA m'interpelle vivement. À titre d'illustration, les crédits engagés en faveur des biens immeubles, productifs de revenus dans les bâtiments publics, dont les mairies, les écoles ou les terrains sportifs, n'entrent plus dans le champ de compensation du FCTVA. Il s'agit pourtant de dépenses engagées au nom de l'intérêt général en faveur d'édifices structurants dans le quotidien de nos concitoyens habitant dans les territoires les plus ruraux. Quelles mesures le Gouvernement prendra-t-il pour renforcer la stabilité dans la durée de la liste des dépenses éligibles et favoriser la prévision des dépenses pour nos élus ?

automatisation a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était définie par des critères juridiques. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate en fonction de leur imputation comptable sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel modifié du 30 décembre 2020. Le périmètre des comptes du plan comptable des collectivités ne permet pas de faire coïncider exactement l'assiette automatisée et l'assiette réglementaire précédant la réforme.

qui enregistre les dépenses relatives aux immeubles privés productifs de revenus, sont inéligibles au bénéfice du fonds. Malgré l'exclusion de ce compte, une part significative des dépenses relatives aux bâtiments privés a néanmoins été rendue éligible, notamment le compte « Constructions en cours ». Cet effet d'assiette est restreint, dans la mesure où les dépenses relatives à la construction de bâtiments publics, parmi lesquels les mairies et les écoles, sont pleinement éligibles. S'agissant des agencements et aménagements de terrains, certains comptes n'ont pas été retenus dans l'assiette automatisée, car ils comportent des dépenses hors taxe, par nature inéligibles au FCTVA., d'autres dépenses auparavant inéligibles ont été rendues éligibles, principalement les dépenses relatives à des biens mis à disposition de tiers. Je rappelle que ce fonds demeure, par principe, un soutien global de l'État en faveur de l'investissement local et ne peut être assimilé à une subvention ou à un concours attribué spécifiquement

et numérique. Madame la ministre, ma question concerne la délocalisation de l'usine Latécoère implantée sur la zone d'activités de Montredon, à Toulouse. Inaugurée voilà à peine cinq ans, et qualifiée alors d'« usine du futur », celle-ci n'abritera plus aucun emploi industriel fin 2024. C'est ce qu'a annoncé, début février 2023, la direction de ce groupe historiquement toulousain, mais dont l'actionnaire majoritaire est aujourd'hui Searchlight Capital Partners, un fonds d'investissement américain. Les machines ultramodernes du site de Montredon, sur lesquelles travaillent encore aujourd'hui 110 personnes, vont quant à elles s'envoler vers les sites à bas coût du groupe en République tchèque et au Mexique. inquiétons bien évidemment en priorité de l'avenir des salariés de ce site, mais cette délocalisation soulève également d'autres questions. Ainsi, en 2016 et 2017, alors que le groupe Latécoère, faute de solution immobilière, menaçait déjà de quitter l'agglomération toulousaine, Toulouse Métropole l'avait assisté dans sa recherche de foncier. En parallèle, Latécoère a bénéficié du programme stratégique de l'État baptisé « Usine du futur », recevant à ce titre 5,4 millions d'euros, ainsi que près de 800 000 euros de fonds européens gérés et versés par la région Occitanie. Les expériences malheureuses se multiplient. La région toulousaine, qui a déjà connu pareilles déconvenues récemment dans le secteur des microconducteurs ou de l'industrie pharmaceutique, n'est pas un cas isolé dans notre pays. Aussi, madame la ministre, l'État pourrait-il envisager de mettre en oeuvre des mécanismes de remboursement de ces aides publiques ou des délais d'engagement lorsque les objectifs affichés de développement de l'activité et de créations d'emplois ne sont manifestement pas visés ou atteints à terme ?

en cas de fraude ou, au titre de l'article L. 773-2 du code de commerce, lorsque le tribunal constate qu'une entreprise de plus de 1 000 salariés n'a pas respecté ses obligations légales de recherche d'un repreneur. Dans ce cas, les personnes publiques peuvent, dans un délai d'un an à compter de ce jugement, demander remboursement de tout ou partie des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi attribuées à l'entreprise au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture.

dans le cadre de nos priorités industrielles stratégiques. Elles sont conditionnées à la réalisation effective de l'investissement et nous sommes attentifs au maintien en France des équipements financés.

du plan France Relance au titre des actions de soutien au secteur aéronautique pour un projet multi-sites. Nous regrettons vivement la décision prise par l'entreprise concernant le site de Toulouse-Montredon et lui avons clairement fait savoir.

En l'état, les défaillances encore constatées aujourd'hui affectent la création d'entreprises artisanales, menaçant jusqu'à l'existence même du secteur des métiers et de l'artisanat,

Un système complexe et peu lisible rend la reconnaissance de la nature artisanale de l'activité particulièrement difficile. La qualité et la précision du registre national des entreprises, conçu pour regrouper les données

de l'activité et de la qualification artisanales ? Le réseau des CMA a formulé des propositions à la mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de

Depuis son ouverture, il y a eu 500 000 formalités enregistrées sur les outils guichet unique et guichet entreprise, dont 300 000 créations et 200 000 modifications et cessations. Concernant les difficultés spécifiques du secteur de l'artisanat, que vous avez

porte sur le périmètre retenu dans le décret d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 2023. Celui-ci doit en effet fixer la liste des nouvelles communes relevant du dispositif « zones tendues ». Sur de nombreux territoires touristiques, de montagne et littoraux, de jeunes ménages se retrouvent dans l'impossibilité de se loger face à la concurrence de nouveaux arrivants disposant d'un pouvoir d'achat très important. Cet engouement résidentiel, accentué par la crise sanitaire du covid-19 et le développement du télétravail, entraîne plusieurs effets pervers et provoque des déséquilibres importants au sein de nos communes : inaccessibilité des logements, réduction de la population sédentarisée, vieillissement de la population, fermetures d'école, phénomènes de surpopulation en période estivale ou encore difficultés de recrutement pour les entreprises. Forte de ce constat, ma collègue Nadège Havet a alerté le Gouvernement ces derniers mois afin de trouver des solutions concrètes pour nos communes.

Désormais, là où existent des difficultés sérieuses d'accès au logement du fait du prix du marché et d'une proportion élevée de logements non affectés à l'habitation principale, de nouveaux territoires vont pouvoir entrer dans le décret dit des zones tendues, et appliquer la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires dès 2024. Nous soutenons pleinement cette avancée. En effet, loin de représenter une pression une pression fiscale supplémentaire s'imposant à l'ensemble des Français, l'élargissement de ce dispositif fiscal, qui restera à la discrétion des maires, est de nature à dégager des marges de manoeuvre pour les collectivités concernées. Le décret, qui répond à une forte demande de nombreux élus- nous pensons en particulier aux élus insulaires -, ne sera cependant une réponse satisfaisante qu'à la condition qu'il soit suffisamment large. Aussi, nous souhaiterions avoir des précisions sur les critères retenus pour arrêter la liste des communes éligibles, ainsi que sur le calendrier d'application de cette mesure très attendue. La

La première concerne l'élargissement du zonage de la taxe sur les logements vacants (TLV) et de la majoration facultative de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS). La seconde a pour objet l'augmentation des taux de TLV, portés respectivement à 17 % la première année et à 34 % à compter de la deuxième, contre respectivement 12,5 % et 25 %. Avant ces modifications, le dispositif zones tendues ne concernait que les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements,

l'est Mme Havet, porte cette question. C'est la raison pour laquelle le zonage intègre désormais des communes, qui, sans appartenir à une zone d'agglomération de plus de 50 000 habitants, présentent une forte tension immobilière. En même temps que les critères relatifs aux niveaux élevés des loyers

particulièrement confrontées à des difficultés spécifiques d'accès à l'habitation principale. Enfin, je vous précise que le décret d'application procédant à la mise à jour de la liste des communes où ces dispositifs sont applicables fait actuellement l'objet,

Le rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) sur la protection sociale des travailleurs indépendants de septembre 2020 a confirmé que, à revenu égal, un travailleur indépendant paie plus de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) qu'un salarié. Afin de réduire l'iniquité entre indépendants et par rapport aux salariés, ce même rapport a préconisé une réforme de l'assiette de cotisations. Selon le Haut Conseil, un abattement forfaitaire de 30 % permettrait d'assurer un traitement équitable entre travailleurs indépendants et salariés. Si un tel abattement figurait bien à l'article 21 du projet de réforme des retraites présenté en 2019, il n'a pas été repris dans le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le dossier de presse du projet de loi soulignait cependant la nécessité de « parvenir à une équité contributive entre les salariés et les indépendants en précisant qu'une concertation serait engagée avec les représentants des différentes professions concernées et leurs organismes de sécurité sociale. Madame la ministre, pouvez-vous confirmer les intentions du Gouvernement à ce sujet ? Faudra-t-il attendre la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ? La parole

le rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale de septembre 2020 a permis de souligner certains travers du système de prélèvements sociaux concernant les travailleurs indépendants.

de 2021. En outre, plusieurs baisses des prélèvements sont intervenues et ont permis, depuis 2015, de réduire de 35 % à 26,5 % le taux global de cotisations applicable aux revenus les plus faibles, en intégrant notamment la baisse de 550 euros 550 euros par an au niveau du Smic intervenue depuis la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022. Le constat d'une complexité des prélèvements sociaux des indépendants demeure particulier, le calcul des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée est circulaire, ce qui le rend difficilement lisible- c'est un euphémisme -pour les travailleurs concernés. concernés. Les assiettes sur lesquelles sont fondés ces calculs, différentes pour les cotisations et la CSG-CRDS, mais aussi distinctes de celle des salariés, défavorisent la formation de droits contributifs, et notamment de droits à retraite, pour les indépendants. C'est pourquoi le Gouvernement a pris l'engagement, dans le cadre de la réforme des retraites, d'engager le chantier de la réforme de l'assiette sociale des indépendants, afin d'en simplifier drastiquement les modalités de calcul, à prélèvements globaux constants.

concerne les pouvoirs attentatoires aux libertés individuelles et à la vie privée de leurs clients qui sont accordés aux banques. La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme doit incomber aux pouvoirs publics et non pas à des organismes privés. Si les banques ont des soupçons, elles doivent alerter la police et les services fiscaux, mais certainement pas se comporter comme une véritable « gestapo privée », en étant autorisées à exercer sur leurs clients des pressions exorbitantes.

Les banques sont des établissements financiers assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, au titre de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. Elles sont ainsi tenues de mettre en oeuvre des mesures dites de vigilance, qui consistent à identifier leurs clients, à vérifier leur identité, à recueillir des informations sur l'objet et la nature de leur relation d'affaires avec eux et à mettre à jour ces informations L'article R. 561-12 du code monétaire et financier prévoit en outre que « la nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires ». Un arrêté pris en 2009 énumère de manière exhaustive les informations susceptibles d'être recueillies pendant toute la durée de la relation d'affaires aux fins d'évaluation de ces risques. Il s'agit surtout d'informations permettant d'évaluer la situation économique, financière et professionnelle du client, ainsi que l'origine et la destination des fonds. En principe, conformément à ce que la loi prévoit, les banques sont tenues de faire part à leurs clients des raisons qui les poussent à leur demander ces informations de l'utilisation qui en sera faite. Elles doivent également informer les clients des conséquences qu'entraîne un refus de leur part de fournir les informations demandées. Chaque banque détermine librement les modalités et dispositifs internes par lesquels elle

Les banques sont enfin tenues de déclarer à Tracfin, la cellule de renseignement financier rattachée au ministère de l'économie, « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ». En tant que détectrices de premier niveau des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, les banques procèdent donc aux signalements nécessaires

hausse des prix de l'énergie, dépendance aux énergies fossiles, part significative de réacteurs des centrales nucléaires à l'arrêt en début d'hiver dernier ... C'est dans ce contexte que le Gouvernement a proposé au Parlement d'étudier successivement deux textes, l'un sur le développement des énergies renouvelables et l'autre sur la relance de l'énergie nucléaire. Ils sont tous deux les bienvenus. Le constat qui s'impose à nous avec une très grande gravité est que l'Union européenne n'est plus en mesure d'assurer sa souveraineté énergétique. Notre continent paie aujourd'hui au prix fort un aveuglement inouï sur ce sujet. Quand certains pays, parmi nos plus proches alliés, ont fait le choix délibéré du gaz et du charbon russes, tout en fermant leurs capacités de production nucléaires en parfait état de fonctionnement, on aurait pu qualifier cette décision de « but contre son camp de « but contre son camp ». En dépit des critiques sur le modèle énergétique français, ce dernier apparaît plus que jamais exemplaire en matière d'empreinte environnementale et d'indépendance énergétique. Il revient donc au Gouvernement, ainsi qu'à la représentation nationale, d'en faire la promotion active sur la scène européenne.

Madame la ministre, ma question est simple. Pouvez-vous, devant la représentation sénatoriale, faire le point sur les objectifs futurs de cette alliance ainsi que sur les prochaines échéances importantes permettant de

Ces deux premières réunions ont été l'occasion de construire un programme de travail commun, autour des questions d'innovation, de recherche et développement, de chaînes de valeur, de compétences, de sûreté de gestion des déchets ou encore d'indépendance vis-à-vis des approvisionnements russes. L'écosystème européen en matière de nucléaire est riche. Nous devons nous appuyer dessus pour mener à bien

indispensable pour la stabilité du réseau européen. Les deux premières réunions de ce groupe de coopération du nucléaire ont permis d'affirmer conjointement le besoin d'un cadre juridique et financier

En effet, pour le seul secteur de la maison individuelle, l'abandon des chaudières engendrerait une pointe estimée à 15 gigawatts supplémentaires, soit l'équivalent de neuf EPR () ; cela suppose qu'elles soient remplacées par des pompes à chaleur performantes. Dans le secteur du logement collectif, il n'existe aucune solution technique autre que les radiateurs électriques pour remplacer les chaudières individuelles. Le changement de source d'énergie pour le chauffage n'est pas l'élément premier de la transition écologique. Il est impératif d'accélérer la rénovation thermique pour diviser par cinq la consommation en kilowattheure par mètre carré, quelle que soit la source d'énergie. Cette décision entraînerait également des conséquences économiques importantes. En effet, les chaudières sont majoritairement produites en France et en Allemagne, à la différence des pompes à chaleur, dont la valeur de marché se situe pour moitié en Asie. Il est entendu que la décarbonation des utilisations du gaz dans les bâtiments doit être une priorité. Néanmoins, une mesure d'interdiction des chaudières serait contre-productive et affecterait le développement du gaz renouvelable, en limitant à terme la capacité d'intégration de ces gaz verts dans les réseaux, ou obligerait à recourir à des systèmes coûteux de rebours vers les réseaux de transport et de stockage. Plutôt que d'interdire les chaudières, il conviendrait de renforcer le soutien au développement de la méthanisation, en s'appuyant sur un modèle agricole résilient et durable et en favorisant notamment les boucles locales de consommation.

imposer le recours à une part importante d'énergie décarbonée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans les logements neufs. Cette première échéance a été imposée aux maisons individuelles. Elle sera progressivement étendue aux logements collectifs en 2025 et aux bâtiments tertiaires. Son objet est de poursuivre l'amélioration de la performance énergétique

est vieillissant, et la construction de nouveaux EPR, dont les coûts sont considérables, ne se feront pas au détriment du développement des énergies renouvelables, pour lesquelles la France est le mauvais élève européen

un délégué interministériel au nouveau nucléaire été nommé pour coordonner ce programme et veiller au respect des délais, des coûts et des niveaux de qualité attendus.

prendra toutes les prescriptions qu'elle jugera nécessaires pour garantir la sécurité de notre parc nucléaire. Ainsi, la ministre Agnès Pannier-Runacher poursuit la stratégie énergétique, et énergique !, du Gouvernement,

Depuis les premières difficultés énergétiques et les conséquences de l'inflation sur les matières premières ou sur les ressources de nos concitoyens, nos artisans vacillent. Et chaque difficulté supplémentaire les fragilise un peu plus. Or, depuis le 1 janvier 2023, les formalités auxquelles sont soumis les artisans et les entreprises sont régies par un guichet unique dématérialisé

Ce guichet unique, rappelons-le, s'appuie sur le registre national des entreprises, qui se substitue aux trois registres nationaux existants : le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers, ainsi que le registre des actifs agricoles.

à responsabilité limitée (EIRL), indispensable pour les entreprises en grande difficulté, n'était à ce jour pas possible, de même que l'inscription des personnes mariées sous le régime de la séparation. Les frais de greffe sont aléatoirement justifiés ou non à l'échelle du territoire. Enfin, les chambres de métiers et de l'artisanat se trouvent dans l'impossibilité de fournir des extraits d'inscription issus du registre national des entreprises. La synthèse obtenue à l'issue de la validation n'est reconnue ni par les banques, ni par les assureurs,

et d'expertise nationale va être diligentée pour accompagner les évolutions de la réponse à Autun. L'ARS s'est ainsi engagée dans un travail de coconstruction de solutions avec l'ensemble des partenaires. Aussi, elle a proposé de créer une maternité territoriale « Saône-et-Loire Nièvre » pour offrir une réponse sécurisée et coordonnée, et des centres de

au motif qu'ils ont failli à l'obligation de repos en exerçant leurs fonctions électives, alors que cette activité n'est pas autorisée explicitement par leur médecin et ne figure pas sur leur arrêt de travail. Cette situation est d'autant plus ubuesque lorsque l'arrêt de travail autorise à l'élu des sorties libres

De plus, il semblerait souhaitable que les élus locaux en arrêt de travail ne soient plus pénalisés dans de telles circonstances, alors qu'ils ont le courage de poursuivre leur mandat malgré la maladie. L'exercice d'un mandat municipal, notamment dans les plus petites communes, exige une forme de continuité du service public difficilement compatible avec une quelconque interruption d'activité. Il serait donc souhaitable que la CPAM fasse preuve d'une certaine clémence à l'égard de ceux qui s'investissent sans compter pour la collectivité publique et d'une certaine forme de discernement selon les cas. Ainsi, il ne semble pas sérieux de considérer qu'un élu en arrêt de travail pour une jambe cassée mette son obligation de repos en péril en participant à une séance du conseil municipal

(Cnam) participe aux campagnes de sensibilisation sur le sujet. Elle a ainsi actualisé sa communication en rappelant, au sein de la rubrique du site de l'assurance maladie consacrée aux élus locaux, la protection sociale qui leur est accordée, notamment leur droit aux indemnités journalières en cas de maladie.

Dans le premier cas, il est bien indiqué que l'élu en arrêt maladie continue à percevoir ses indemnités journalières au titre de son incapacité de travailler s'il continue à exercer son mandat local dans le cadre de l'autorisation donnée par le médecin prescripteur.

d'arrêt de travail. Celui-ci comprend l'ajout d'une mention spécialement réservée aux élus locaux pour rappeler très clairement aux médecins qu'ils peuvent les autoriser à exercer leur activité au titre du mandat électif pendant l'arrêt maladie.

Les travaux techniques ont abouti récemment ; le nouveau formulaire sera disponible prochainement.

Dans un contexte de pénurie de médecins en zone rurale et de fortes inégalités territoriales, ces structures sont nécessaires à l'équilibre global de l'offre médicale. Or la Croix-Rouge semble s'employer à les fermer méthodiquement.

par la Croix-Rouge. Ces centres sont des structures déclarées auprès de l'ARS, mais ne bénéficient ni d'autorisations ni de financements spécifiques, qui permettraient à celle-ci d'influer sur les décisions des organismes gestionnaires.

Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, un comité de pilotage national de suivi a été mis en place en janvier 2022. En Haute-Vienne, les sept CSI sont déficitaires. La Croix-Rouge en a déjà fermé trois, au motif de problématiques de recrutement. Pour les quatre autres, la Croix-Rouge serait à la recherche de repreneurs, mais sans perspective à ce jour. Pour le CSI d'Ambazac, les infirmières actuellement salariées envisagent de reprendre elles-mêmes l'activité, et elles étudient la forme juridique la plus adaptée. Le directeur du développement de la Croix-Rouge française a assuré à l'ARS qu'en l'absence de solutions de reprise, la Croix-Rouge maintiendrait l'activité des CSI. Aucun engagement écrit n'a toutefois été transmis en ce sens. Si l'ARS ne peut s'opposer à la fermeture de centres de santé, il est nécessaire de travailler localement à une fluidification de la communication et du partage d'information de la Croix-Rouge, afin que les ARS, et en l'occurrence celle de Nouvelle-Aquitaine, puissent anticiper des solutions de poursuite des prises en charge. Plus globalement, le ministère a conscience des difficultés financières rencontrées par les CSI et du besoin de réinterroger leur modèle économique. À ce titre, le Gouvernement a annoncé en février dernier le versement d'une aide exceptionnelle de 11 millions d'euros en 2023 aux CSI régis par la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile

Dans le cas de Ruffec, nous avons obtenu très récemment un sursis grâce à l'arrivée, la semaine dernière, d'un médecin intérimaire. Ce recrutement opportun permettra de maintenir les vingt-neuf lits menacés et d'éviter la fermeture du service de médecine polyvalente. Mais cela ne change pas la situation sur le long terme. pour exemple le centre hospitalier d'Angoulême, qui a dû fermer son service d'angioplastie le week-end du fait d'un manque de médecins intérimaires. L'intérim est devenu pour bon nombre d'hôpitaux un mal nécessaire,

épargne les cliniques privées, qui sont pourtant en tête des rémunérations pour les pays de l'OCDE. Le Ségur de la santé a malheureusement oublié la permanence des soins et la pénibilité. La loi Rist, entre en application ce mois-ci, n'a pas été suffisamment anticipée. Pire, vous combattez l'intérim avant d'avoir restauré l'attractivité des carrières hospitalières. Votre annonce, bienvenue, de la semaine dernière relative à la revalorisation de 20 % du plafond pour les intérimaires et à la prime de solidarité territoriale (PST) démontre votre impréparation lorsqu'il s'agit de penser l'accès aux soins dans nos territoires ruraux. Vous savez l'ensemble des élus locaux mobilisés pour l'aide à l'installation de praticiens. Quelles mesures prévoyez-vous de mettre en place pour soutenir nos hôpitaux de proximité, comme celui de Ruffec, et pour prévenir des risques de fermeture de services dans nos territoires ?

face aux tensions actuelles sur la démographie des professionnels du soin, le centre hospitalier de Ruffec fait face à d'importantes difficultés et doit périodiquement ajuster son fonctionnement à la réalité des personnels présents, avec des réductions de capacités dans les services de médecine ou de Dans ce contexte, afin de maintenir la continuité des soins, l'établissement est amené à faire appel à des remplaçants intérimaires pour fonctionner. Le centre hospitalier de Ruffec présente une dégradation de ses résultats financiers due à une baisse d'activité et à des charges majorées, du fait notamment de ce recours à l'intérim. Cet intérim médical, par ailleurs, pour protéger les hôpitaux, est plafonné dans ses montants depuis hier, date d'entrée en application de la loi Rist- vous l'avez souligné. L'ARS accompagne avec la plus grande attention l'hôpital de Ruffec, qui a ainsi pu bénéficier de mesures de soutien 1,127 million d'euros au titre de la restauration des marges financières de l'établissement ; 674 000 euros supplémentaires pour soutenir l'hôpital, soit un total de 1,8 million d'euros, qui fait l'objet d'une dotation sur dix ans. L'arrivée d'une nouvelle direction pour les centres hospitaliers d'Angoulême, de La Rochefoucauld et de Ruffec permettra également d'impulser une dynamique de solidarité territoriale et de consolidation de l'hôpital de Ruffec dans son environnement, en lien avec les autres établissements du territoire, en s'appuyant sur de réels atouts

Un travail est également engagé sur l'attractivité médicale autour de projets nouveaux, en lien avec le service de médecine : développement d'hospitalisations de jour ; création de postes partagés entre le centre hospitalier d'Angoulême et celui de Ruffec. Par ailleurs, à court terme, une solution un contrat de remplacement a été trouvée pour permettre la continuité de fonctionnement du service de médecine du centre hospitalier de Ruffec pour le mois d'avril, et les équipes du centre hospitalier en lien avec l'ARS recherchent des solutions pérennes.

personnes handicapées. Je souhaite attirer une nouvelle fois votre attention, madame la ministre, sur les dispositifs Ségur et ceux qui sont issus de la mission sur les métiers de l'autonomie. En effet, les services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad), relevant de la compétence des départements, sont exclus de ces dispositifs, alors qu'ils rencontrent des difficultés de recrutement susceptibles de mettre en péril ce service tout à fait essentiel. L'aide de la qui prend la forme d'une participation fixée par décret à 50 % des financements versés par les départements, dans la limite de 200 millions d'euros par an, ne suffit pas à répondre aux enjeux financiers au regard de son niveau, mais aussi du non-cumul avec le bénéfice de l'avenant 43 et du Ségur. dès lors, une inégalité de traitement incompréhensible entre les salariés exerçant au sein d'établissements et ceux des services sociaux et médico-sociaux exerçant à domicile. J'élargis ma question, tant les difficultés et les incompréhensions sont croissantes s'agissant de ceux qu'il est désormais convenu d'appeler les « exclus du Ségur », aux établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Alors qu'il avait été souligné au moment de l'épidémie de covid-19 que chaque membre de l'équipe, quelle que soit sa mission, assurait un lien essentiel avec l'usager, il semble que cela soit aujourd'hui oublié- pourtant, un projet d'établissement concerne tout le monde.

Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser mon collègue Jean-Christophe Combe, qui m'a demandé de répondre à votre question. L'État, aux côtés des départements, a pris d'ores et déjà des décisions historiques en augmentant de 4 milliards d'euros les rémunérations des professionnels du secteur social et médico-social. Au total, ce sont près de 700 000 salariés qui ont bénéficié d'une revalorisation de 183 euros net mensuels, dont environ 500 000 au titre du Ségur et de la mission dite Laforcade, et 200 000 à la suite des annonces de la Conférence des métiers du 18 février 2022. Il est évidemment nécessaire de poursuivre les efforts et les mesures à destination de l'ensemble des professionnels pour contribuer à l'amélioration de la qualité et de l'accompagnement, des conditions de travail, des parcours, et plus largement pour favoriser leur valorisation. Le renforcement de l'attractivité du secteur passera par une transformation profonde des parcours professionnels et des voies d'accès aux métiers sociaux et médico-sociaux. Le Gouvernement est pleinement engagé en ce sens. Afin d'attirer tous les talents et de valoriser l'expérience acquise, nous engageons, avec le ministre du travail, une réforme profonde des dispositifs de validation des acquis de l'expérience (VAE). Nous soutenons également le développement massif de l'apprentissage. Nous adaptons les formations initiales et continues pour répondre aux évolutions des métiers. Enfin, nous mobilisons les acteurs du service public de l'emploi pour permettre l'orientation et les reconversions des demandeurs d'emploi. J'ajoute que, pour les agents de la fonction publique concernés, le projet de refonte des carrières et rémunérations de la fonction publique, annoncé par mon collègue Stanislas Guerini, permettra de répondre à ces différents enjeux et d'assurer une refonte de la grille indiciaire de certains professionnels. par ailleurs, aux côtés des représentants des employeurs et des salariés, appelé à la construction d'une convention collective unique pour le secteur social et médico-social. Depuis le 18 février 2022, le Gouvernement plaide pour avancer sur ce sujet dans le cadre du dialogue social. C'est la condition d'une revalorisation durable des parcours professionnels de l'ensemble des personnels du secteur, y compris techniques et administratifs. Je rappelle que l'État et l'Assemblée des départements de France (ADF) ont annoncé, le 18 février 2022, qu'ils étaient prêts à mobiliser 500 millions d'euros pour faire aboutir ces travaux.

Dans le contexte de crise sanitaire que nous avons connu, et en réponse à l'immense mobilisation des personnels d'accompagnement des personnes fragiles durant cette période, le Gouvernement a accordé successivement à certaines catégories professionnelles la prime dite Ségur, d'un montant de 183 euros. Ces décisions ont permis de souligner la reconnaissance nationale pour les efforts considérables fournis et de revaloriser des professions dont l'attractivité a beaucoup diminué ces dernières années. Toutefois, bien des frustrations ont été ressenties par les personnels exclus du bénéfice de cette prime : certains professionnels de services sociaux et de prévention en santé- par exemple, les infirmiers qui instruisent les demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) -et nombre de professions administratives, techniques et logistiques du secteur social et médico-social. Les conséquences de ces inégalités

J'évoquais, en réponse à votre collègue Stéphane Sautarel, les augmentations à hauteur de 4 milliards d'euros des rémunérations des professionnels du secteur social et médico-social. C'est un effort important, mais vous avez raison de souligner qu'il nous faut poursuivre les efforts, notamment pour mieux valoriser ces professionnels, en travaillant sur la question salariale, bien sûr, mais pas seulement. d'exemple, le Gouvernement, en lien avec les fédérations d'aide à domicile, a consacré la journée du 17 mars dernier aux aides à domicile, pour leur dire merci et valoriser ce métier, essentiel aujourd'hui, et qui le sera encore davantage demain. L'amélioration de l'attractivité de notre secteur passera donc par une transformation profonde des parcours professionnels et des voies d'accès aux métiers sociaux et médico-sociaux, en refondant les dispositifs de VAE, en soutenant l'apprentissage et en adaptant les formations. En outre, pour les agents de la fonction publique concernés, le projet de refonte des carrières et des rémunérations de la fonction publique, que mon collègue Stanislas Guerini a annoncé, permettra de répondre à ces différents enjeux et d'assurer une refonte de la grille indiciaire de certains professionnels. Enfin, je le redis, nous avons, aux côtés des représentants des employeurs et des salariés, appelé à la construction d'une convention collective unique pour le secteur social et médico-social. C'est la condition d'une revalorisation durable des parcours professionnels de l'ensemble des personnels du secteur, y compris techniques techniques et administratifs. L'État et l'Assemblée des départements de France ont annoncé, le 18 février 2022, qu'ils étaient prêts à mobiliser 500 millions d'euros pour faire aboutir ces travaux. Nous sommes convaincus que les discussions relatives à l'augmentation des rémunérations, notamment les plus bas salaires, doivent pleinement prendre leur place dans le cadre cette convention collective unique étendue.

toujours relogés dans des chambres doubles au centre hospitalier de Limoux, qui lui-même est en situation de gestion de crise. Pourtant, je me souviens des mots adressés par le ministre Christophe Castaner aux Audois, deux jours après la catastrophe : « L'État participera afin que tous les équipements publics arrachés à votre terre soient reconstruits. » Dans l'Aude, madame la ministre, nous n'avons pas la mémoire courte ! Ces mots apparaissent comme une promesse non tenue, car, manifestement, le provisoire dure toujours, et avec lui la souffrance de ces patients déracinés de leur foyer d'accueil. Pire, ce retard à un coût, évalué à 10 millions d'euros en 2019. Le projet de reconstruction est resté, hélas ! à l'état de pré-étude opérationnelle. Plus on tarde et plus le coût de reconstruction explose : c'est 20 millions d'euros qu'il faut aujourd'hui prévoir. J'ose espérer qu'il n'y a pas

Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur, dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, le département de l'Aude a effectivement vécu un dramatique épisode méditerranéen. Cette inondation a entraîné l'évacuation de l'Ehpad de Saint-Hilaire, d'une capacité de 52 places, et les dégâts ont nécessité sa reconstruction un projet estimé à 10 millions d'euros en 2019. Le bâtiment de l'Ehpad n'était en effet plus exploitable au regard du caractère persistant du risque inondation. La solution temporaire retenue par les autorités a été la délocalisation des places de l'Ehpad dans quatre sites relevant du centre hospitalier de Limoux, avec le maintien des emplois. Dès 2018, plus de 1 million d'euros étaient alloués à l'Ehpad par l'ARS Occitanie, et chaque acteur concerné partageait l'importance de définir rapidement un projet de reconstruction afin de permettre l'exploitation de l'intégralité de la capacité autorisée et d'accompagner les personnes accueillies. Ainsi, plusieurs mesures financières et d'octroi de dispositifs supplémentaires aux 52 places d'hébergement permanent ont été anticipées. D'une part, le conseil départemental de l'Aude a autorisé l'agrément de 10 places de résidence autonomie. D'autre part, l'ARS Occitanie a prévu une subvention d'investissement de 2,1 millions d'euros inscrite dans le cadre du Ségur de l'investissement, mais également : un pôle d'activités et de soins adaptés de 14 places permettant d'améliorer la prise en charge des personnes souffrant de maladies neurodégénératives ; 6 places d'accueil de jour ; 2 places d'hébergement temporaire. Monsieur le sénateur, comme vous le soulignez, le dernier projet présenté par le centre hospitalier de Limoux n'est pas satisfaisant. De son niveau de financement découlerait un prix de journée qui serait inaccessible pour la population de la commune, ce qui n'est évidemment pas acceptable. Je sais que la direction du centre est en lien avec les autorités de tutelle afin de présenter un projet de reconstruction cohérent, qui soit ouvert et inscrit dans la vie de la commune de Saint-Hilaire.

Madame la ministre, les structures collectives de garde de la petite enfance à Paris, notamment les crèches associatives ou municipales, proposent une offre d'accueil indispensable pour la plupart des familles de la capitale. Depuis plusieurs années, une pénurie de places disponibles est constatée dans ces établissements. Dans certains arrondissements, la Ville de Paris indique même que les commissions d'attribution des places en crèche ne peuvent attribuer plus de 40 % des places initialement ouvertes, faute d'auxiliaires de puériculture récemment diplômés : 1 047 postes seraient toujours vacants, avec pour conséquence la fermeture de 3 680 places. Cette situation risque de mettre en grande difficulté de très nombreuses familles parisiennes. J'aimerais donc savoir, madame la ministre, au-delà de la campagne sur les métiers de la petite enfance déjà promise par la Première ministre, ce que le Gouvernement faire pour assurer une revalorisation et une promotion des métiers de la petite enfance, et connaître le calendrier de validation des diplômes qui permettrait à la Ville de Paris et aux structures privées de procéder à des recrutements pour envisager les prochaines rentrées dans des conditions plus normales. Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice, le Gouvernement porte une attention particulière au secteur de la petite enfance, qui souffre de problèmes structurels liés à la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et aux besoins croissants des familles. L'enjeu est celui des crèches collectives, mais pas seulement. Car le vieillissement des assistantes maternelles actuellement en poste est aussi un enjeu majeur. des allocations familiales (Cnaf), 10 000 professionnels manquent aujourd'hui à l'appel sur l'ensemble du territoire et le nombre de places offertes par les assistants maternels recule en raison de départs massifs à la retraite. En conséquence, ce sont plus de 160 000 parents qui sont empêchés de prendre ou de reprendre un emploi, faute de mode d'accueil adapté à leurs besoins et à leurs moyens. Cela concerne bien sûr la ville de Paris, au même titre que le reste du territoire. ambition est d'accroître massivement le nombre de places, avec 200 000 places d'accueil supplémentaires qui devront être créées à horizon 2030. Cet objectif quantitatif se double bien sûr d'un objectif qualitatif, et les deux sont pleinement liés, car la qualité d'accueil repose en grande partie sur un nombre de professionnels formés, en nombre suffisant. C'est toute l'ambition du service public de la petite enfance, et c'est pour y répondre que nous avons engagé un travail partenarial avec les acteurs, dans le cadre du comité de filière Petite enfance. Car cette ambition ne pourra se concrétiser sans un travail en profondeur sur la formation et les parcours, les conditions de travail et la rémunération des professionnels de la petite enfance. En outre, mon collègue Jean-Christophe Combe a souhaité lancer une campagne ambitieuse de promotion de l'ensemble des métiers de la petite enfance. Cette campagne, visible à partir de la mi-avril, permettra de découvrir toute la richesse et l'importance de ces métiers de sens qui requièrent connaissances et compétences spécifiques. Il faut évoquer aussi les travaux de préfiguration de l'observatoire national de la qualité de vie au travail (ONQVT), qui se poursuivent. En parallèle, une mission a été confiée à l'Igas pour animer les travaux de définition du socle social commun des professionnels de la petite enfance, contrepartie demandée aux partenaires sociaux pour la participation de l'État au financement de revalorisations dans le secteur. Beaucoup d'autres actions sont en cours, par exemple sur les formations, toutes sous-tendues par l'idée d'atteindre le plus vite possible nos objectifs.